Républicains. L'annonce d'une possible cession de l'entreprise Saint-Gobain basée à Pont-à-Mousson à son concurrent chinois a fait l'effet d'une bombe, d'abord pour les 2 000 salariés lorrains de l'entreprise. effet un vrai coup de tonnerre, car il s'agit du premier employeur privé du bassin d'emploi du sud du département de Meurthe-et-Moselle, fort de plus de 500 000 habitants. Alors que le Gouvernement affiche à l'envi sa volonté de conduire une politique industrielle ambitieuse et conquérante, comment entend-il garantir le maintien sous pavillon français de tous nos brevets, consacrant ainsi la très haute valeur ajoutée du savoir-faire français, mondialement connu, avec Saint-Gobain ? Par ailleurs, pour cette activité sensible, comment entend-il protéger et garantir nos intérêts stratégiques dans la mondialisation ? cette entreprise ne lutte pas à armes égales, en raison de normes sociales et environnementales particulièrement exigeantes auxquelles échappent ses concurrents. Quand donc vous mobiliserez-vous avec l'Union européenne pour exiger la réciprocité normative pour les investissements étrangers en France ?

Le groupe a annoncé aux représentants du personnel avoir ouvert une réflexion autour de la recherche de partenariats au mois de février dernier. Vous connaissez la situation mieux que quiconque : depuis la crise de 2008, les commandes de canalisations à l'entreprise de Pont-à-Mousson ont été divisées par deux. Des concurrents chinois et indiens ont émergé, faisant perdre à ce site de nombreuses parts de marché, notamment dans les pays du Golfe. Un projet de compétitivité visant à concentrer des investissements et des activités sur le site de Pont-à-Mousson a été engagé, avec 133 millions d'euros d'investissements dans les quatre ans dans les quatre ans qui viennent. En outre, un transfert de production d'Allemagne vers la France se traduit notamment par la relocalisation de quatre-vingts emplois. Telle est la situation actuelle. Ces efforts, certes nécessaires, ne sont pas suffisants pour renforcer durablement le site de Pont-à-Mousson. Saint-Gobain n'exclut pas d'ouvrir le capital de sa filiale.

qui se trouveraient sacrifiés sur l'autel d'une mondialisation aveugle et destructrice, où tous ne jouent pas à armes égales. Nous avons besoin de plus de France et de mieux d'Europe.

Cela commence avec l'inspiration catastrophique du Premier ministre de l'époque, David Cameron, qui souhaitait se relégitimer à bon compte grâce à un référendum gagné d'avance, un peu comme un footballeur qui dribblerait le poteau de pour On sait ce qu'il est advenu : un réveil avec une gueule de bois, un peuple britannique qui a été victime des menteurs et des populistes et le « non » qui l'a emporté de peu. C'est d'ailleurs une leçon à méditer pour tous les gouvernements en quête de légitimité. Le mauvais feuilleton se poursuit au parlement britannique et à la Chambre des communes. Débat après débat, vote après vote, les parlementaires britanniques montrent le triste spectacle de ceux qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent Face à ces turbulences subies par le gouvernement et le parlement britanniques, il est essentiel que l'Union européenne montre un visage d'unité, de solidité et de sérénité. C'est ce à quoi s'est exercé avec conviction et savoir-faire Michel Barnier. Les populistes se sont trouvés sans voix Aujourd'hui, les Britanniques demandent un nouveau délai. Nous le comprenons, parce que nous voulons éviter le Brexit. Mais quel est le sens de la décision du Conseil européen d'accorder un délai supplémentaire au gouvernement britannique ? Est-ce pour rouvrir la négociation ou pour laisser du temps au parlement britannique pour voter l'accord négocié ? Quelle réponse pouvons-nous apporter aux entreprises et aux personnes concernées pour les rassurer et leur permettre d'exercer sereinement leur activité ? La parole

Il s'agit non pas de rouvrir les négociations de l'accord de retrait, mais de laisser aux autorités britanniques le temps de procéder à sa ratification en permettant un retrait ordonné. De la même manière, les conclusions du Conseil européen de cette nuit précisent que le délai supplémentaire ne peut pas être utilisé pour rouvrir les négociations sur les relations futures. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous sommes disposés à amender la déclaration politique sur les relations futures si la position britannique venait à évoluer. Mais la négociation des modalités de celles-ci ne s'ouvrira qu'après le retrait du Royaume-Uni. Vous le voyez, le calendrier est établi. Un délai supplémentaire est accordé. Mais il appartient désormais aux Britanniques de déterminer s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne dans les termes convenus dans l'accord,

Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part. » La parole

accordé au Royaume-Uni un nouveau délai, jusqu'au 31 octobre prochain, pour permettre au parlement britannique de ratifier l'accord de retrait déjà maintes fois rejeté par cette instance. Il faut dont a fait preuve la France quant à la durée du nouveau délai a permis de conjurer l'impasse institutionnelle et politique qui aurait pu survenir si celui-ci s'était étendu au-delà de la date d'installation de la future commission européenne, fixée au 1 novembre prochain. Nous ne pouvons que nous en féliciter. L'Union européenne et ses futures instances ont tant de défis à relever que nous ne pouvons clairement pas nous permettre d'affronter un éventuel blocage de son fonctionnement.

très vraisemblablement à participer aux élections européennes le 23 mai prochain. Nous y verrons un peu plus clair, au Royaume-Uni comme dans le reste

Mais, cette nuit, la France a été entendue et l'Union européenne a été préservée. Une extension trop longue aurait pu être comprise comme la volonté de l'Union de retarder ou d'annuler le Brexit. Nous devons respecter le choix souverain du peuple britannique. C'était notre première priorité. Le Conseil européen a donc décidé d'accorder une extension jusqu'au 31 octobre. À cette date, la page du Brexit aura été tournée, et la nouvelle commission européenne pourra prendre ses fonctions le 1 novembre en se consacrant pleinement à ses travaux, à son ambition et aux projets concrets, au bénéfice des citoyens européens. Notre deuxième priorité était de ne était de ne pas décider à la place des Britanniques. Il leur appartient de choisir d'organiser ou non des élections européennes : s'ils ne le font pas, ils quitteront l'Union le 1 juin ; s'ils le font, les parlementaires britanniques élus quitteront le Parlement européen lorsque le Royaume-Uni sortira Enfin, et c'est évidemment le plus important pour nous, la troisième priorité était de préserver le fonctionnement de l'Union. Londres devra donc s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril les objectifs européens. Mme May s'y est engagée par écrit, et le Conseil européen l'a redit très clairement. Vous avez raison, monsieur le sénateur : nous devons veiller avec le Conseil européen, qui fera un point en juin, à examiner très attentivement le respect par le Royaume-Uni de ses engagements. Vous le voyez, nous voulons- Jean-Yves Le Drian l'a rappelé -un retrait ordonné. Mais nous sommes prêts à tous les scénarios. Je serai demain à Calais et à Boulogne-sur-Mer pour rencontrer nos concitoyens qui vivent de la pêche et qui seraient en première ligne en cas d'absence d'accord.

Dans son avis du 4 avril dernier, l'Autorité de la concurrence recommande d'élargir la vente des médicaments sans ordonnance à la grande distribution. Cela ne peut que réjouir l'un des principaux leaders, qui annonce depuis des années à quel point il fera baisser les prix des médicaments dans l'intérêt du consommateur.

Dans certains cas, ils peuvent avoir des effets secondaires très graves. Les pharmaciens d'officine assurent une mission de santé publique au service des 4 millions de Français qui entrent chaque jour dans une pharmacie. Dans les zones fragiles, ils assurent souvent seuls l'accès aux soins et un service de garde jour et nuit, ce que ne fera certainement pas la grande distribution. Ils ont un rôle irremplaçable de conseil

sous une apparence bénigne, le paracétamol est toxique à des posologies peu supérieures aux doses thérapeutiques. Malgré les dispositions de votre projet de loi sur la santé, madame la ministre, il n'y aura pas d'amélioration concernant la désertification médicale avant dix ans. Permettre la vente de médicaments dans les grandes surfaces fragiliserait financièrement les officines et remettrait gravement en cause le maillage territorial des pharmacies, stratégique en matière d'accès à la santé sur l'ensemble du territoire national, en particulier en zone rurale. En 2018, tous les trois jours,

; j'espère que nous aiderons à présent les démocrates soudanais à réussir une transition civile. Cela dit, la réélection de Benyamin Netanyahou menace comme jamais l'avenir d'une solution de paix entre Israël et les Palestiniens. À la tête d'une nouvelle coalition d'extrême droite, il veut désormais annexer la Cisjordanie occupée. Avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, une colonisation galopante, le feu vert américain à l'annexion du Golan, Netanyahou et Trump piétinent sans vergogne les résolutions de l'ONU et veulent enterrer cette fois la solution à deux États. Leur projet déboucherait sur un seul État discriminatoire et colonial, réduisant 6,5 millions de Palestiniens à vivre sans droits, sans État, parqués derrière un mur de la honte. Je reviens d'Israël et des territoires palestiniens où je me suis rendu en compagnie d'une quarantaine d'élus locaux français. La situation est terrible Tous les Palestiniens, ceux d'Israël, comme ceux de Jérusalem, de Cisjordanie et de Gaza, sont discriminés, chassés par les colons, empêchés de vivre, de travailler et de circuler. Avec 700 et des incursions meurtrières quotidiennes, près de 300 colonies ou avant-postes, un mur de 700 kilomètres qui a coûté la destruction de 400 000 oliviers, leur vie est un enfer.

Benyamin Netanyahou est adoubé par les extrêmes droites européennes. Notre inertie ressemble de plus en plus à une capitulation. Il faut conclure ! Monsieur le ministre, la voix de la France doit se faire entendre avec force et courage dans ce moment crucial. Allez-vous enfin reconnaître l'État de Palestine pour dire clairement « stop » au processus d'annexion ? La France va-t-elle enfin agir pour des sanctions internationales contre un gouvernement qui bafoue si gravement les droits humains et le droit international ?

que nous suivons avec beaucoup d'attention. Nous souhaitons que le départ de M. el-Béchir puisse ouvrir la voie à une solution pacifique.

Je ne voudrais pas faire de commentaire particulier. D'abord, les résultats n'ont pas encore été proclamés officiellement, même s'il apparaît que l'issue du vote est claire et que le parti du Premier ministre Netanyahou et ses alliés sont sortis vainqueurs du scrutin, puisque leur principal adversaire, M. Gantz, l'a reconnu hier.

aide à l'Unrwa pour compenser le retrait américain. Je vous remercie de le reconnaître. La position de la France n'a pas changé. Nous sommes attachés à un cadre : le droit international, avec les résolutions du Conseil de sécurité auxquelles vous faites référence.

socialiste et républicain. J'habite depuis toujours à douze kilomètres des fonderies de Pont-à-Mousson, qui tournent depuis plus de 150 ans. Elles font partie de notre identité et sont une fierté collective, d'abord pour les 2 000 salariés du groupe et leur savoir-faire mondialement reconnu, puisque l'on trouve partout les canalisations en fonte ductile et les fameuses plaques d'égout. Or Saint-Gobain s'apprête à lâcher le fleuron Pont-à-Mousson vous venez de nous confirmer que la cession était possible, mais aussi que la filière relevait bien d'une activité pouvant être considérée comme stratégique. Vous venez aussi de nous dire que vous nous recevrez après votre rendez-vous avec le PDG du groupe Saint-Gobain et qu'alors seulement, vous nous donnerez plus d'informations. Je vous remercie de nous rencontrer de manière unitaire, mais je suis le quatrième parlementaire à vous interroger sur le sujet cette semaine, et votre réponse demeure insatisfaisante. Car c'est bien vous qui définissez la politique industrielle de la France. Je vous demande donc quelles sont vos lignes rouges et claires sur ce dossier, en amont de ce rendez-vous. Quelles informations quant à la santé financière du groupe Saint-Gobain justifiant qu'il se sépare du site de Pont-à-Mousson avez-vous ? Par ailleurs, vous disposez de leviers, ici et avec les fonds européens, pour contribuer à une modernisation et éviter une délocalisation désastreuse pour notre économie, pour l'emploi, pour le pays, et empêcher ainsi la perte des brevets et des savoir-faire historiques de la fonderie. La Lorraine a déjà beaucoup trop payé pour la désindustrialisation. Merci de nous rassurer

Nous parlons de la situation d'un site qui vient de bénéficier d'un engagement d'investissement de plus de 100 millions d'euros et qui est en train de recruter quatre-vingts emplois supplémentaires. Je pense donc qu'il faut replacer le sujet dans son juste positionnement. Il est question d'une possible ouverture de capital,

c'est l'un des derniers sites de production de canalisations en Europe. C'est probablement un atout, de même que la présence de savoir-faire anciens et d'un certain nombre d'avances technologiques par rapport aux concurrents indiens et chinois. C'est tout l'enjeu de la discussion qui va s'ouvrir maintenant

qui engage peut-on bâtir pour préserver l'emploi ? Il faut conclure ! Nous ne voulons pas d'un accord capitalistique avec les Chinois ou d'autres qui dépouillerait les salariés, le territoire et la France.

79 % de la totalité des sapeurs-pompiers. Il est inutile de souligner combien leur action est capitale pour la santé et la sécurité, en particulier dans le monde rural.

du fait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les sapeurs-pompiers volontaires seraient désormais considérés non plus comme des citoyens librement engagés au service de nos compatriotes, mais comme des travailleurs à part entière, avec toutes les conséquences juridiques, sociales et économiques qui en découlent. En un mot, ce serait la fin d'une organisation que la loi française a consacrée en donnant un cadre juridique adapté aux sapeurs-pompiers volontaires par la loi du 20 juillet 2011, adoptée à l'unanimité par le Parlement.

Sénat a appelé la Commission et le Parlement européen à adopter une directive spécifique pour protéger le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Le maintien de leur statut n'est pas seulement l'expression d'une vision altruiste et exemplaire, il est aussi la base sur laquelle reposent les services d'incendie et de secours de nos départements. Je rappelle que, en milieu rural, 100 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires qui interviennent, certes pour combattre les incendies, mais

vous êtes au courant puisque votre assemblée a saisi la Commission européenne à ce sujet -de travailler au niveau européen. Peut-on modifier la directive de 2003 ? Faut-il lancer une nouvelle initiative ? Nous sommes prêts à accompagner une démarche en ce sens visant à donner un cadre protecteur à l'ensemble des engagements citoyens,

au Brexit. Je m'exprime également au nom du président Cambon, qui est retenu aujourd'hui au Mali auprès de nos soldats français. Nous sommes tous deux particulièrement inquiets de l'évolution du dossier du Brexit depuis bientôt trois ans

ne sait pas, quand et comment sortir de l'Union. Cette décision géostratégique funeste a été prise par un peuple aujourd'hui désorienté, que l'on a hier trompé, suite d'un référendum décidé par l'ancien Premier ministre David Cameron, lequel n'a rien trouvé de mieux que de prendre l'Europe tout entière en otage pour régler un problème intérieur ! Monsieur le ministre, Bruxelles a pris hier la décision de prolonger une nouvelle fois la date de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Ma question est simple : pourquoi une telle décision et comment contrôler la sincérité et l'attitude des soixante-treize parlementaires britanniques de nouveau présents demain au Parlement européen, à une période particulièrement critique où il faudra voter sur le nouveau cadre financier pluriannuel et, surtout, décider de la nouvelle composition de la Commission et désigner

La décision qui a été prise cette nuit permet de respecter quatre principes fondamentaux pour nous tous : les intérêts de l'Union européenne ; le vote démocratique britannique

31 000 d'entre eux ont été touchés par des effets invalidants dus à la prise de leur nouveau traitement, sans qu'ils bénéficient de la moindre écoute de la part de leur médecin traitant ou de votre ministère, qui se rangeaient derrière l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament Une récente étude franco-britannique démontre clairement que les deux versions du traitement commercialisé par l'entreprise Merck n'étaient pas forcément substituables.

lorsqu'il est absorbé, induit des différences de dosage chez les patients, individuellement. Cette étude ne remet pas en cause l'étude antérieure qui avait conclu à l'équivalence de biodisponibilité. Elle souligne simplement qu'il s'agit d'un médicament auquel chaque individu a une sensibilité très différente. Cela peut expliquer l'ensemble des effets

je vous remercie

La semaine prochaine, des petits-déjeuners gratuits seront proposés dans huit académies tests. Ces mesures étaient attendues depuis longtemps dans les zones où se concentrent les populations les plus défavorisées. Monsieur le ministre, l'école de la République doit redevenir un facteur de justice sociale et permettre l'égalité des chances. Je salue donc ces dispositions de bon sens qui s'attaquent aux racines des inégalités et complètent les mesures phares que sont le dédoublement des classes de CP et de CE1 ou celles que vous défendrez sur ce banc dans quelques semaines : la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans ; la visite médicale obligatoire pour les enfants entre 3 et 4 ans. S'attaquer aux inégalités à la source est le nerf de la guerre, afin de favoriser l'égalité des chances pour plus de justice sociale.

Rappelons également que la sous-alimentation en France, qui certes reste faible, à un taux d'environ 3 %, n'a pas régressé depuis vingt ans. Un élève qui n'a rien avalé le matin ne produira pas les efforts intellectuels nécessaires à un apprentissage efficace. Monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur les différentes mesures que vous avez déjà mises en place pour assurer une meilleure justice sociale et poursuivre votre engagement en ce sens ? sens ? Avez-vous un calendrier précis relatif à l'élargissement du dispositif « cantine à un euro » à tout le territoire ?

Ce résultat est essentiel, comme j'ai eu souvent l'occasion de le vérifier dans mes précédentes fonctions. Nous devons évidemment faire en sorte que les enfants soient bien nourris si nous voulons qu'ils apprennent correctement, de même que nous devons veiller à leur santé.

est le partenaire des collectivités locales. Nous allons aider les municipalités à réaliser ce qu'elles font déjà ou ce qu'elles voudront faire en la matière. Autrement dit, pour les communes, notamment celles

du ministre de l'intérieur, je veux aujourd'hui vous parler de Luciano, artiste de reggae jamaïcain mondialement connu. Comme moi, Luciano vient de cette belle et grande région, la Caraïbe, qui fit autrefois la richesse des puissantes métropoles. Une communauté de nations de plus de 40 millions d'habitants qui tente depuis quelques années de poser les bases d'une coopération solide. Luciano et ses musiciens devaient venir en Martinique pour un concert très attendu, le 31 mars dernier. Mais ce jour-là, le concert n'a pas eu lieu : les musiciens n'ont pas obtenu leurs visas dans les temps.

Depuis un peu plus d'un an, nos voisins jamaïcains et la plupart des ressortissants des grandes Antilles doivent passer par le consulat général de Washington pour venir chez nous. Comme bien d'autres consulats, celui de Washington a confié le traitement des demandes de visas à un prestataire privé, tristement dénommé VFS. Ce prestataire privé, qui coûte cher à ceux qui veulent venir chez nous, ne répond ni aux mails ni aux appels téléphoniques, et ne permet pas de suivre correctement les demandes. Il décourage les visiteurs et tue à petit feu toute tentative de coopération ou d'échanges économiques, culturels ou touristiques. Faciliter la délivrance de visas pour des courts séjours dans notre territoire ne provoquera pas, je vous rassure, un afflux massif de Jamaïcains en Martinique ! Et notre territoire ne fait pas partie de l'espace Schengen. Les postures coloniales ont tout fait pour nous faire tourner le dos à ce bassin légitime, cette « géographie cordiale » si bien nommée par le poète. Le chemin inverse est long et compliqué. Mon pays a tout mis en oeuvre, parfois à marche forcée, pour intégrer les grandes instances caribéennes. Il est désormais membre de l'Association des États

d'une manière générale, sur l'attractivité des départements et collectivités d'outre-mer au travers de la dispense de visas pour les ressortissants étrangers.

à la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet arrêté prévoit d'ores et déjà un certain nombre de dispenses à la possession d'un visa de court séjour pour

mobiles. C'est le cas à Kingston, où un prestataire envoie les demandes à notre consulat général à Washington. Généralement, les demandes sont traitées très rapidement.

et qui sont aujourd'hui injustement, pour ne pas dire scandaleusement, présentés comme des nantis. Les choix que vous avez faits jusqu'ici sont clairs : les retraités sont les boucs émissaires du nouveau monde. Vous avez décidé sciemment de baisser leur pouvoir d'achat en désindexant les retraites et en augmentant la contribution Depuis votre arrivée au pouvoir, les retraités-avec les classes moyennes-sont les grands perdants de votre politique. Ils ont perdu près de 400 euros par an et par ménage. Alors que les études publiées récemment montrent que le pouvoir d'achat des retraités ne cesse de décroître, vous faites entendre une petite musique : les retraités en France sont trop riches, trop aisés, trop privilégiés.

retraite en France est élevé. C'est oublier que la vertu de notre modèle social est justement de permettre à nos anciens de vivre décemment. CGT ! Madame la ministre, la réforme des retraites s'annonce et l'heure des choix approche. Allez-vous persister dans la direction que vous avez choisie depuis le début du quinquennat, à savoir la déconstruction de notre modèle social et la paupérisation de tous les retraités ? Ou allez-vous proposer une réforme qui respecte ceux qui ont toujours eu droit à une retraite sereine ? J'ai cru comprendre que vous hésitiez sur le chemin à suivre. Votre question ! Les retraités manifestent aujourd'hui leur mécontentement. Madame la ministre, éclairez-nous

jour, une mesure qui entrera en vigueur avant la fin de l'année. Nous avons mis en place le 100 % santé, qui permettra de couvrir complètement les frais d'optique, de prothèses dentaires et d'audioprothèses. Il entrera en vigueur dès cette année pour les prothèses auditives et dentaires. Nous avons fait le choix de revaloriser drastiquement le minimum vieillesse en l'augmentant de 100 euros en deux ans et demi : il atteindra 903 euros au 1 janvier prochain. C'est la plus grande revalorisation du minimum vieillesse lancée ces dernières années,

Ces performances, nous ne les avions pas vues depuis bien longtemps. Nous baissons les impôts et les cotisations salariales, et je ne reviendrai pas sur les nombreuses mesures prises en la matière, notamment la suppression de la taxe d'habitation,

Ce programme de stabilité a été établi avant l'annonce des décisions de sortie du grand débat, mais, comme vous le savez, en la matière, nous prendrons des décisions qui s'inscriront dans l'objectif de soutenabilité de nos comptes publics. Je veux dire le lien entre ce pacte de stabilité et le programme national de réformes que nous menons. Ce programme vise, en premier lieu, à refonder notre modèle social pour construire une société plus juste. Les mesures structurelles que nous avons prises en matière de formation, d'apprentissage et de réforme du marché du travail, ainsi que les mesures d'urgence sociale

de mensonges ... Nous regrettons ce grand décalage entre les shows, les annonces, voire les forfanteries, et la réalité vécue par les Français.

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 3,

que nous transmettions systématiquement les procès-verbaux des infractions relatives à la chasse aux fédérations départementales des chasseurs, la commission est allée plus loin en prévoyant également la transmission systématique

de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS. Conformément à sa mission de préservation et de restauration de la biodiversité, l'office français de la biodiversité et de la chasse conventionnera avec la Fédération nationale des chasseurs pour que le réseau des fédérations des chasseurs mette en oeuvre des actions définies par cette convention. La FNC propose notamment des actions relatives à la restauration de la nature ordinaire et de la trame écologique, à la préservation des espaces protégés, à la préservation des espèces chassables et protégées, à la connaissance des écosystèmes, des espèces et des populations.

ce fonds soit « alimenté par le financement mentionné au troisième alinéa », relatif au permis de chasse national, et que « l'État ou ses établissements publics apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier pour un montant de 10 euros par permis de chasser national validé dans l'année à la réalisation des actions mentionnées

par cohérence avec les modifications apportées par les amendements n 209 rectifié et 210 rectifié. Il s'agit en particulier de maintenir une contribution de l'État aux actions des fédérations à hauteur de 10 euros par permis départemental, le fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs.

qui comprend, d'une part, une section d'indemnisation des dégâts de grand gibier et, d'autre part, une section de péréquation, destinée à atténuer les écarts entre fédérations départementales en matière de ressources et de charges. Or certaines fédérations, comme celle du Territoire de Belfort, font face à des déséquilibres structurels entre leurs ressources et leurs besoins de financement. Je le sais, la le sais, la Fédération nationale a prévu de mettre en place un dispositif de soutien aux fédérations en difficulté qui permettrait d'examiner, au cas par cas, la situation des fédérations, et de leur apporter un soutien si nécessaire. Néanmoins, il s'agit d'un engagement, qui n'a pas la même force qu'une disposition juridique. Compte tenu de ces éléments, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat. Quel est l'avis du Gouvernement ?

un appui financier. Cet amendement vise à établir un droit, pour une fédération départementale, à obtenir une aide la Fédération nationale, ce qui va à l'encontre de l'objectif de responsabilisation des fédérations départementales.

d'opposition à l'intégration de terrains dans le territoire d'une ACCA en vue de préserver le périmètre de ces associations, dont la mise en place répond à un objectif de regroupement et de meilleure gestion des territoires de chasse.

souligné lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement comprend le souhait de garantir la stabilité dans le temps des territoires des associations communales de chasse agréées, même si la rédaction des dispositions concernées peut soulever des questions juridiques au regard du respect du droit de propriété. Le

Autant les réserves de chasse sont utiles pour permettre un renouvellement du petit gibier, voire pour le préserver et le gérer au mieux, autant elles font souvent obstacle à une régulation efficace du grand gibier.

Lever l'obligation de constituer une réserve de chasse pour le grand gibier est donc un vrai facteur de simplification pour la régulation du gibier. En cela, ces deux amendements identiques me paraissent fortement utiles. Le sous-amendement vise à maintenir la faculté de créer une réserve pour le grand gibier lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

les ACCA favorisent, sur leur territoire, le développement de gibier, de la faune sauvage, dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique et la régulation des nuisibles.

Seules les ACCA sont soumises à ces obligations de réserve.

Cet amendement vise à mentionner expressément la possibilité pour l'autorité administrative d'imposer le prélèvement d'animaux dans un délai déterminé, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

En outre, l'article L. 425-5-1 permet déjà au préfet de notifier à un détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné, avec ensuite la possibilité d'engager

celui des titres permanents, qui sera géré par l'OFBC, et celui des validations et autorisations de chasser, qui restera géré par la Fédération nationale des chasseurs. Par ailleurs, le dispositif proposé précise les modalités de transmission et d'actualisation des données par les fédérations départementales et par le gestionnaire de chaque fichier central. Les modifications proposées permettent de préciser et de préserver le rôle de la FNC, qui ne se verra pas dépossédée de tout rôle en la matière, à la différence du dispositif du projet de loi initial, qui avait suscité des craintes de la part du monde de la chasse. La commission est donc favorable

par la fédération départementale des chasseurs visant à prévenir la diffusion des dangers sanitaires et à assurer la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, l'adoption de ces amendements permettra d'éviter les dérives conduisant aujourd'hui à fragmenter certains territoires. La commission a donc émis un avis favorable sur ces amendements

rapporteur. Nous souhaitons également lutter contre l'engrillagement des espaces naturels et forestiers, afin de mieux prévenir les risques sanitaires et les atteintes à la continuité écologique. L'adoption de ces amendements y contribuerait en renforçant l'encadrement de la gestion à l'intérieur des enclos.

l'amendement n° 169. Depuis plusieurs années, sur de nombreux territoires, les chasseurs sont confrontés à une raréfaction du petit gibier de plaine- lièvres, cailles, perdrix, faisans ... -, ce qui implique parfois des plans de gestion draconiens avec une limitation, voire une interdiction, de prélèvements de ces espèces dans les territoires concernés. Pour compenser, les chasseurs effectuent en conséquence de nombreux relâchers. Or, en l'absence de recensement et de contrôle réglementaire, aucune estimation précise n'existe quant aux quantités d'animaux d'élevages relâchés dans le milieu naturel. Aucun chiffre viable n'existe, faute de contrôle. Selon les sources- éleveurs de petit gibier ou associations de protection de la nature -les estimations oscillent entre 10 millions et 30 millions de spécimens relâchés chaque année, en France, dans le seul but de maintenir une activité de chasse de petit gibier.

Pour remédier à cet angle mort dans notre droit, cet amendement vise à modifier l'article L. 424-11 du code l'environnement pour élargir le dispositif de recensement et de contrôle des prélèvements et relâchers de grand gibier et de lapins à toutes les espèces relâchées. Nous souhaitons réellement

à renforcer les actions collectives de prévention, en fixant des règles nationales de sécurité pour la chasse collective à tir de grand gibier qui soient valables et homogènes dans tous les départements, et en instaurant, dans chaque fédération départementale, une commission de sécurité à la chasse. tend à généraliser des règles qui sont déjà mises en oeuvre dans de nombreuses fédérations départementales et qui ciblent les actions de battue au grand gibier, les plus accidentogènes. Il s'agit en particulier de généraliser le port d'effets fluorescents- pratique déjà en vigueur dans la plupart des départements de signaler ses actions à proximité des voies publiques, puisque le gibier peut traverser les voies, et de prévoir la remise à niveau par le biais d'une formation obligatoire tous les dix ans aux bonnes pratiques de sécurité.

pris par le ministre chargé de la chasse, après concertation avec la Fédération nationale des chasseurs. En outre, une commission départementale de sécurité de la chasse sera mise en place au sein de chaque fédération départementale ; c'est une bonne solution. Au terme

le nourrissage consiste à fournir un apport à des animaux à des périodes sensibles où la disponibilité alimentaire dans les milieux et les habitats naturels ne s'avère pas suffisante. L'agrainage, c'est donner à manger tout le temps.

détermineront les conditions et les localisations de l'agrainage dissuasif, en fonction des départements et des périodes de l'année.

Je me félicite que les chasseurs aient fini par prendre la mesure des dégâts causés par la multiplication anarchique des sangliers, notamment en termes d'impact sur l'activité agricole. Ainsi, à cause de l'égrainage, de l'élevage illégal et d'une gestion inadaptée, les sangliers sont passés dans le pays de quelques dizaines de milliers d'individus dans les années 1960 à plus d'un million au XXI siècle. Ils sont responsables de 80 % des dégâts déclarés, pour un coût de plus de 50 millions d'euros. Cette multiplication a entraîné une explosion des nuisances : dégâts sur les cultures, dégâts dans nos communes et accidents de la route se chiffrant à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les chasseurs sont dépassés et n'arrivent plus à réguler cette population, comme en témoigne cet amendement, qui émane des représentants des chasseurs. Il faut naturellement interdire l'agrainage. Nous étions même tentés de ne permettre aucune exception. Temporairement, pour ne pas aggraver la situation de nos agriculteurs, nous vous proposons néanmoins une rédaction qui prévoit comme seule exception à cette interdiction la protection des cultures.

est défavorable à cet amendement, qui tend à établir une relation déséquilibrée entre les documents cynégétiques et les documents de gestion forestière, en donnant un caractère automatique à l'établissement d'un plan de chasse visant à atteindre les objectifs fixés dans les documents d'aménagement des forêts, qui relèvent eux-mêmes du régime forestier.

? En prévoyant une consultation des communes forestières, cet amendement permet de renforcer la prise en compte des questions sylvicole lors de l'élaboration des plans de chasse, sans imposer de contraintes excessives au monde cynégétique. C'est une évolution utile, eu égard à l'impact du grand gibier sur certains peuplements forestiers. Cela fera

introduit en commission. Celui-ci tend à instaurer une procédure particulière pour l'élaboration des plans de chasse communaux pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, tout en précisant que « les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en oeuvre du plan de chasse ». La notion d'« organisations représentatives des communes » ne semble pas suffisamment précise. La représentativité d'une organisation de collectivités n'étant pas définie, une telle rédaction risque de multiplier de façon trop importante le nombre d'organisations sollicitées pour avis avis avant la mise en oeuvre des plans de chasse. Ainsi, le présent amendement tend à solliciter l'avis de la seule Association départementale des maires,

Selon les territoires concernés, l'une ou l'autre des rédactions proposées pourra être plus appropriée. Dès lors qu'il s'agit d'une question très précise liée aux spécificités du régime de droit local en Alsace-Moselle, nous avons souhaité nous en remettre à l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il me semble que, tout au long de ces débats, vous nous avez demandé de faire confiance au terrain, de nous adapter aux spécificités locales et de ne pas tout définir trop précisément. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement. La formulation adoptée en commission évoque la consultation des organisations représentatives des communes et donne donc plus de souplesse pour consulter de matière adaptée ces communes

de la direction départementale des territoires à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Je comprends cette mesure, car on ne peut pas demander à longueur d'année la diminution du nombre des fonctionnaires et ne pas en accepter les conséquences pratiques. en Alsace-Moselle, les communes adjugent la chasse tous les ans « au nom et pour le compte des propriétaires fonciers ». Le plan de chasse, c'est-à-dire le nombre de bracelets attribués à chaque lot de chasse et les dégâts des cervidés sont un élément déterminant de la valeur cynégétique et, finalement, Il est donc normal que les communes soient consultées par la fédération des chasseurs. Je remercie la commission d'avoir inscrit une telle disposition dans le projet de loi et adopté la rédaction que je lui avais proposée. Cette dernière a été imaginée par l'Institut de droit local alsacien-mosellan, pour tenir compte des réalités dans les trois départements concernés. Selon un proverbe alsacien, le diable se cache dans les détails. de l'amendement n° 58 rectifié illustrent parfaitement ! En effet, la question est de savoir à qui les présidents des fédérations des chasseurs doivent écrire pour désigner leurs interlocuteurs. En Alsace, ces présidents vous répondront spontanément, tout comme le préfet d'ailleurs, qu'ils écriront au président de l'association départementale des maires et au président de l'association des communes forestières d'Alsace, sachant que ces deux personnes se concertent régulièrement. En Moselle, le président de la fédération des chasseurs vous répondra spontanément, comme le préfet d'ailleurs, qu'il écrira à l'Association des communes rurales. En effet, l'association départementale des maires ne s'intéresse pas aux questions relatives ce destinataire le comité des communes forestières de la région du Grand Est. Les trois présidents des trois fédérations de chasseurs et les trois préfets savent donc très bien quelles sont « les organisations représentatives des communes En conséquence, c'est la rédaction retenue par la commission qui est la bonne.

complémentaires concernant la fixation des prélèvements des espèces de grands gibiers, que ce soit en plus ou en moins, pour être sûr de ne pas se tromper.

François Patriat. Le transfert de la gestion des plans de chasse individuels aux fédérations départementales des chasseurs vise à mieux les responsabiliser- ils le demandent, et c'est une bonne chose -, pour maîtriser les populations de grand gibier et les dégâts que celles-ci suscitent, l'État fixant les objectifs de résultats sans déterminer dans le détail les moyens pour atteindre ces objectifs. L'État détermine les objectifs, mais les moyens restent à la charge des fédérations. Cet amendement vise à ne pas trop atténuer la responsabilisation des chasseurs, en cantonnant l'intervention de l'État aux seules situations où elle est nécessaire.

afin de lui permettre de demander une modification dans un nombre plus diversifié de situations et, en particulier, en cas d'augmentation des dégâts de gibier. En outre, ces dispositions que la fixation des quotas de prélèvement sera faite à une échelle territoriale suffisamment fine, pour mieux lutter contre les dégâts des espèces soumises à un plan de chasse. Il s'agit d'un signal très fort en faveur des agriculteurs et des forestiers. L'adoption de cet amendement remettrait en cause les avancées obtenues en commission. La commission émet

dans les cas strictement nécessaires. Il s'agit de ne pas trop atténuer la responsabilisation des chasseurs.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à compléter les dispositions actuelles, qui se limitent à la prise en compte des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique,

il semble important que le préfet, dans le cadre de son arbitrage, puisse prendre en compte les conclusions de la commission régionale sylvo-cynégétique à laquelle, je le rappelle, les chasseurs participent.

par une commission essentiellement compétente en matière de forêt, sauf à rompre les équilibres existant entre ces deux activités. En outre, les plans de chasse individuels sont aussi soumis, je le rappelle, au schéma départemental de gestion cynégétique, qui doit lui-même être compatible avec le programme régional de la

il n'apparaît pas clairement que la gestion adaptative proposée ne concernera que les espèces chassables. Le concept de gestion adaptative, qui n'a pas de fondement juridique ou scientifique, pourrait donc s'appliquer à toutes les espèces, y compris les Pourtant, aux termes du droit de l'Union européenne, les espèces protégées ne sont pas chassables. Elles ne peuvent être régulées que dans des conditions dérogatoires cumulatives très strictes. Il nous semble donc impératif de préciser clairement que cette notion ne s'appliquera qu'aux espèces chassables. Quel est l'avis de la commission ? Les espèces

En tout état de cause, la gestion adaptative ne saurait conduire à remettre en cause la protection des espèces qui s'impose, en application du droit européen. La commission émet donc un avis

Cardoux, pour explication de vote.

l'amendement n° 112. L'Assemblée nationale a intégré dans le projet de loi la définition de la gestion adaptative, et je m'en félicite, car c'est l'une des grandes avancées de ce texte. Toutefois, en l'état, le texte ne donne qu'une définition partielle du concept innovant de gestion adaptative. Il s'agit d'être plus précis et plus exhaustif. La gestion adaptative est un changement de logiciel dans la façon dont l'État doit prendre ses décisions, afin de ne pas figer le statut juridique des espèces sauvages- je rejoins sur ce point les propos de Jean-Noël Cardoux.

Au regard de la parfaite connaissance qu'ils ont des différents territoires et des réalités du terrain, leurs retours d'expérience constituent un atout qui doit contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, notamment s'agissant des cormorans

La rédaction actuelle constitue un bon équilibre, dont la mise en oeuvre sera assurée par voie réglementaire. Pour les raisons évoquées à l'instant, il ne nous semble pas opportun de modifier cette rédaction, que ce soit en ajoutant un nouveau qualificatif pour les espèces concernées ou en mentionnant une prise en compte du contexte socio-économique, dont la portée est très imprécise.

à la définition des modalités de mise en oeuvre de la gestion adaptative. Il nous paraît utile de prévoir expressément l'existence de ce dialogue. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le terme

étant déjà incluse dans la définition. En revanche, comme l'a dit M. le rapporteur, il est important de maintenir la référence à l'état de conservation de l'espèce et de son écosystème, pour afficher l'objectif de cette gestion.

Par ailleurs, après avoir été éclairé par ce comité, le ministre soumet toujours sa décision à l'avis des parties prenantes concernées au sein du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Il me semble que cet amendement est donc satisfait.

de la commission ? Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre au sein de la commission. L'identification des espèces relève d'un travail d'expertise qui doit être guidé par une instance indépendante. C'est bien l'objet du comité consultatif d'experts récemment créé en vue d'identifier les espèces pouvant être intégrées à la nouvelle gestion adaptative. Leur identification sera ensuite effectuée par décret. Il ne nous paraît pas opportun de confier l'initiative du processus à la Fédération nationale des chasseurs. Une mise en oeuvre apaisée de la gestion adaptative suppose de ne pas conférer à une partie prenante un poids trop important, au risque de manquer l'objectif visé, à savoir améliorer la gestion de certaines espèces soulevant à ce jour de multiples conflits entre acteurs. La commission émet donc un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis

Mme Anne-Catherine Loisier. Il s'agit de compléter l'assiette de la participation des territoires, afin que celle-ci englobe tous les territoires susceptibles d'influencer le développement des populations de grand gibier, notamment les réserves de chasse, les terrains en opposition à la chasse et les espaces en déshérence cynégétique.

préconisait d'étendre l'assiette de la contribution territoriale aux territoires susceptibles d'être classés. Cela inclut en particulier les réserves de chasse, où cette activité est interdite, ainsi que les terrains qui ont fait l'objet d'un droit d'opposition de la part de leur propriétaire. La commission émet donc un avis défavorable.

Le problème du financement des dégâts occasionnés par le grand gibier est un problème important. Dans certaines fédérations, les montants peuvent être de l'ordre de 400 000 euros ou 500 000 euros, voire davantage. L'effort financier qui est alors demandé aux chasseurs titulaires d'un permis départemental peut donc être très important. Or force est de constater que le chasseur ayant validé un permis de chasse national est dispensé, lui, de s'acquitter de la contribution personnelle instaurée. Nous proposons donc qu'un chasseur qui a validé un permis national soit dans l'obligation de s'acquitter de la participation personnelle demandée pour financer les dégâts de grand gibier. Le chasseur titulaire d'un permis national doit être, nous semble-t-il, solidaire des autres chasseurs s'agissant du financement de ces dégâts. J'ajoute une remarque : le problème, dans certains départements, est que nombre d'associations

chasser, le risque étant d'abandonner les territoires aux sangliers. Dans ces conditions, pourquoi ne pas envisager d'autres solutions de financement, avec un système

au financement des dégâts de grand gibier à hauteur d'un cinquième du montant du permis national de chasser. Ainsi, pour un permis national dont le montant a été réduit, me semble-t-il, à 200 euros par la loi de finances pour 2019, la contribution demandée sera de 40 euros

le rappelle, l'Assemblée nationale a proposé la suppression du timbre national grand gibier, acquitté jusqu'à présent, notre collègue l'a rappelé, par les chasseurs titulaires d'un permis national, en vue d'alimenter le Fonds cynégétique national géré par la FNC et permettant d'aider les fédérations départementales à assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier. La suppression du timbre national grand gibier vise à mettre en oeuvre l'accord conclu entre la FNC

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit à ce titre de généraliser la participation territoriale à l'hectare actuellement mise en place de manière volontaire par certaines fédérations départementales. L'objectif annoncé est de mieux responsabiliser les fédérations en matière de gestion du gibier.

en permettant aux fédérations départementales d'assujettir l'ensemble de leurs adhérents, y compris ceux qui sont dotés d'un permis national, à une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, qui prend parfois la forme d'un timbre départemental. Le droit en vigueur prévoit en effet une dispense de cette participation pour les adhérents titulaires du permis national, en raison du timbre national grand gibier que ces chasseurs acquittent déjà. Dès lors que ces chasseurs n'acquitteront plus ledit timbre, pourquoi continuer à les soustraire à la participation personnelle qui peut être mise en place par une fédération départementale, alors que leurs camarades titulaires d'un permis départemental et adhérents de la même fédération l'acquitteraient ?

quant à la situation des fédérations départementales pour lesquelles une contribution à l'hectare trop élevée risque d'être peu soutenable et de poser, dans certains territoires, La commission a donc collectivement considéré que l'évolution proposée par l'auteur du présent amendement, bien loin de revenir sur la suppression du timbre national, en tire les conséquences logiques et donne des marges de manoeuvre complémentaires aux fédérations locales.

sur ces trois amendements. à l'équilibrer dans des conditions qui ne soient pas insoutenables pour les chasseurs dans certains départements. Par ailleurs, la fédération nationale s'est déjà engagée à soutenir financièrement les fédérations départementales qui en auraient besoin.

François Patriat, pour explication de vote. J'ai à la fois un grand respect pour Roland Courteau et de l'amitié pour lui, et je connais son sens de la justice et de l'équité. Je suis convaincu que l'argument qu'il défend, dans son esprit, est un argument de justice. Reste qu'il

Il y a un problème sur le terrain ; il n'est pas propre à la fédération du département de l'Aude. Je connais d'autres cas, dans d'autres départements.

J'essaie de trouver une solution. M. le rapporteur a bien résumé le fond de ma pensée. Mes chers collègues, je vous parle de solidarité entre les chasseurs titulaires d'un permis national et les chasseurs titulaires d'un permis départemental. Et je ne pense pas

pour sa seule section péréquation, cet amendement vise à sécuriser la situation des seules fédérations départementales des chasseurs à effectifs restreints en demandant à la Fédération nationale des chasseurs de leur apporter une aide

pour présenter l'amendement n° 29 rectifié. Cet amendement a pour objet d'étendre l'opposabilité du schéma départemental de gestion cynégétique aux détenteurs de droit de chasse dans le département, afin que ces mesures soient uniformément applicables sur l'ensemble des territoires où la chasse est pratiquée. cet amendement permettrait aussi de consolider le dispositif prévu pour rendre obligatoire l'instauration par la fédération des chasseurs de la contribution territoriale destinée à sécuriser le financement de la prévention et de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures agricoles.

En outre, ces amendements nous paraissent satisfaits par le droit en vigueur, qui permet déjà d'engager la responsabilité financière d'un détenteur de droit de chasse qui ne procède pas à la régulation des espèces présentes sur son fonds, causant des dégâts de gibier. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements

En conscience, parce que son application a suscité de vives tensions avec les chasseurs et les populations autochtones, qui contestaient sa pleine adaptation au contexte spécifique de la Guyane. La période transitoire qui s'achèvera le 1 janvier 2020 a notamment révélé

auprès des populations de l'intérieur pour constituer, appareil photo en main, des dossiers de permis dans des conditions d'information contestables et l'arrêt prématuré de la vente d'armes de chasse et de cartouches, les services de l'État ont fait preuve d'un empressement et d'une précipitation incompréhensibles, voire incompatibles avec la concertation qu'aurait méritée la mise en place d'un tel dispositif. Une telle mesure ne peut s'imposer d'elle-même au forceps, parce que les services de l'État parce que les services de l'État ont décidé de ne pas s'embarrasser ! Elle aurait nécessité une discussion et l'adhésion de tous. Dans ce contexte, nous, élus- président de collectivité, parlementaires et maires -, nous sommes réunis avec les collectifs de chasseurs à l'occasion des premières assises de la chasse, qui se sont tenues le 1 décembre 2018. Une résolution a été adoptée à l'unanimité, afin de demander, d'une part, un moratoire sur l'application du permis de chasser et, d'autre part, l'élaboration d'un dispositif spécifique à la chasse en Guyane. Cette résolution a été confirmée par un vote, le 10 décembre 2018, de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane. C'est donc conformément à cette résolution que je vous présente cet amendement et que je vous demande d'entendre la voix d'une grande majorité

L'amendement n° 114 rectifié vise, d'une part, à proroger jusqu'en 2023 la période transitoire qui s'achèvera le 1 janvier 2020, et, d'autre part, à supprimer la validation communale existante au profit d'une seule validation départementale annuelle gratuite.

Il s'agit certainement d'une erreur de notre part, mais force est de constater que les premiers permis n'ont été délivrés qu'à partir du 1 janvier 2018. Et si je compte bien, jusqu'au 1 janvier 2020, cela fera deux ans, et non trois ans La logique voudrait donc que l'on proroge d'au moins une année supplémentaire cette période transitoire. Je propose pour ma part d'aller jusqu'en 2023. En effet, je vous l'ai dit, l'application du permis a été particulièrement difficile, compte tenu de l'empressement des services Je pense notamment aux formations qui seront demandées pour l'obtention du permis. Il va sans dire que les populations de l'intérieur ne pourront pas prendre l'avion ou l'hélicoptère pour venir suivre ces formations. Le bon sens voudrait qu'un référent soit présent dans chaque village. Tout cela demande du temps et de la concertation, ce qui nous a toujours manqué dans ce dossier. Enfin, je propose de prévoir la gratuité d'une seule validation départementale annuelle. Le dispositif actuel prévoit une validation communale jugée inadaptée en ce qu'elle limite le périmètre de chasse à deux communes au plus. Non seulement l'échelon communal retenu est inégal en Guyane, puisqu'il existe de fortes disparités entre les communes, mais la chasse guyanaise se caractérise par une grande mobilité, qui ne saurait être limitée dans l'espace, les chasseurs partant parfois plusieurs jours en forêt. De plus, il a été prévu que cette validation communale puisse être gratuite, le maire pouvant fixer à zéro euro le montant de la taxe demandée. Dans ces conditions, je propose de simplifier le dispositif en remplaçant cette validation communale

de chasse vise avant tout à contrôler l'achat et la détention des armes en en faisant le seul moyen d'accès légal aux armes en Guyane. La délivrance du titre de permis de chasser est gratuite jusqu'en 2020 et donnera lieu par la suite à une validation annuelle payante. Si plusieurs associations favorables au permis se sont créées, un collectif d'opposants s'est constitué à l'automne 2017, et en décembre 2018, les élus de la collectivité et les parlementaires ont demandé au Gouvernement un moratoire.

L'instauration du permis de chasser en Guyane vise avant tout à contrôler l'achat et la détention des armes, la détention de ce permis devenant le seul moyen d'accès aux armes. Pour bien contrôler cet accès, tout le dispositif devrait avoir vocation à être déployé dès 2020, avec l'examen préalable à la délivrance du permis et sa validation annuelle, de manière à vérifier que seuls les chasseurs accèdent aux armes. Ce dispositif permet d'interdire la chasse à toute personne interdite d'accès et de détention d'arme. Il est déjà tout à fait spécifique à la Guyane. Ainsi, outre les possibilités de valider un permis au niveau départemental ou au niveau national pour pouvoir chasser sur le territoire correspondant, la loi ÉROM a ouvert la possibilité d'une validation communale. Celle-ci est adaptée aux communes autochtones et à la superficie des communes. Son montant, déterminé par chacune d'entre elles, est plafonné à 22 euros. Les communes où sont majoritairement présentes des communautés pratiquant une chasse traditionnelle de subsistance sont bien évidemment invitées par le Gouvernement à prévoir une validation gratuite, ce qui est tout à fait possible. sa mise en place, en février 2018, le permis de chasse rencontre l'adhésion de la majorité des chasseurs, plus de 5 700 demandes ayant été reçues et 5 300 permis ayant déjà été délivrés sur tout le territoire guyanais. Dès lors, le Gouvernement ne souhaite pas supprimer ou reporter sa mise en place, qui correspond à une avancée importante en matière de contrôle de l'accès aux armes et donc de sûreté publique. Mais il demeure attentif aux éventuelles difficultés que peut susciter la mise en oeuvre de la seconde phase, après 2020. Afin d'améliorer encore le dispositif, notamment pour les populations qui utilisent la chasse comme moyen de subsistance, le Gouvernement est prêt à travailler à une évolution de la loi pour bien rappeler que la validation communale décidée par les maires peut être gratuite et pour permettre aux chasseurs qui le souhaitent de valider leur permis communal pour plus de deux communes limitrophes. Dès lors, le Gouvernement n'est pas favorable à ces trois amendements. La parole est à M.

disposent les petites communes rurales ne leur permettent pas toujours de financer la création d'une police municipale. Cet amendement tend à faire bénéficier aux communes qui souscrivent une convention avec la fédération de chasseurs d'agents de développement chargés d'intervenir pour la régulation de certaines espèces nuisibles, la divagation l'errance des animaux domestiques, la circulation sur les chemins ruraux et la collecte des animaux sauvages morts. Quel est l'avis de la commission ? La

en permettant, sur dérogation, la chasse d'oiseaux migrateurs en dehors des périodes d'ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification. Cet article va par ailleurs plus loin que l'actuel code de l'environnement, en incluant dans la liste des motifs permettant cette dérogation des sujets qui ne sont pas liés à la protection de l'environnement, tels que la sécurité aérienne

nous ne disposerions pas dans notre droit de toutes les marges de manoeuvre permises dans le cadre européen. En outre, je précise que ces dérogations sont rigoureusement encadrées par deux conditions cumulatives : l'absence d'alternative satisfaisante et l'état de bonne conservation des espèces concernées.

pour le ministre chargé de la chasse d'autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective.

Nous l'avons dit-on en introduction de ce débat sur la chasse, le nombre de chasseurs a diminué de moitié en quelques décennies,

Jean-Noël Cardoux et Claude Bérit-Débat, en vue de réaffirmer l'existence des modes de chasse traditionnels. Il s'agit de pratiques spécifiques à certains territoires qui présentent des enjeux culturels très, très, très forts pour ceux-ci.

Nous l'avons gagnée sur les nobles en 1789, et elle fait partie de notre patrimoine commun. Je suis sénateur des Hauts-de-Seine, mais je me rends très souvent en Corrèze ; je mange du gibier ; je participe à des chasses,

Le scrutin est ouvert.

des chasseurs comme gestionnaire d'une réserve naturelle. Cela nous semble cohérent avec la responsabilisation accrue du monde cynégétique en matière de gestion durable de la biodiversité et cela permet de conforter le rôle des fédérations en matière de gestion des espaces naturels. Je précise que le choix du gestionnaire restera à la main du préfet ou du président du conseil régional. En outre, l'encadrement des activités humaines dans une réserve, y compris des activités de chasse, est défini par l'acte de classement, lequel s'impose au gestionnaire. Si la chasse est encadrée, alors cela s'imposera à la fédération concernée.

Mes chers collègues, si vous trouvez cette proposition trop restrictive, je vous invite à voter l'amendement n° 117 rectifié, qui vise à interdire la chasse à tir le mercredi, afin de permettre aux enfants de profiter de la nature et aux chasseurs de pratiquer leur sport, ou leur loisir, favori les jours

Mes chers collègues chasseurs, il me semble que vous serez heureux d'accompagner vos enfants et vos petits-enfants sur les chemins de l'avenir en toute sérénité ! Quel

d'autres territoires à vocation d'accueil du public et où les pouvoirs de police générale du préfet lui permettent, en complément ou en substitution des pouvoirs des maires, de réglementer l'usage des armes à feu lorsque c'est nécessaire. Par ailleurs, nous avons déjà renforcé la sécurité. Le Gouvernement demande

Comme l'a parfaitement rappelé madame la secrétaire d'État, il y a suffisamment d'espaces publics ouverts en France dans lesquels les gens peuvent se promener librement. Je rappelle que, dans les forêts domaniales,

Le scrutin est ouvert.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

afin de tirer les enseignements de retours d'expérience récents. Plus précisément, il s'agit de renforcer le caractère opérationnel et dissuasif des sanctions administratives, notamment en permettant que des mesures conservatoires et de suspension prises par l'autorité administrative à l'égard d'installations, ouvrages ou travaux non autorisés et pouvant porter gravement atteinte à la biodiversité soient assorties d'une astreinte ou d'une exécution d'office. Nous proposons aussi la publication par l'autorité administrative, sur le site internet de l'État dans le département concerné, de l'acte prononçant la sanction administrative, sur le modèle anglo-saxon dit du. Quel est l'avis

avec des associations de protection de la nature. Il y a une méfiance atavique, nous n'allions pas la faire disparaître, comme par enchantement, en quelques jours ... Face à cette méfiance qui demeure,

d'empoigne, si je puis dire, entre ceux de nos collègues qui défendent la Fédération nationale des chasseurs et ceux qui défendent les fédérations départementales de chasseurs. Ainsi, le compromis patiemment bâti depuis des années par tous les acteurs et qui s'est concrétisé à l'Assemblée nationale a été dévoyé, dévoyé, en oubliant que l'intérêt général exige un effort considérable en faveur de la biodiversité, à l'heure où l'humanité est responsable d'une sixième extinction de masse. Dans la discussion par la voix de Guillaume Gontard, nous avions marqué notre attachement à la création de l'OFB, tout en soulignant les faiblesses du texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Le risque demeure que cette fusion soit l'occasion de nouvelles coupes budgétaires, à rebours des ambitions que devrait avoir la France en matière de biodiversité et des promesses du plan biodiversité. La mise à contribution inévitable des agences de l'eau nous inquiète grandement, d'autant que vous avez émis, madame la secrétaire d'État, un avis défavorable sur les amendements tendant à fixer le principe de la préservation des ressources de ces agences. Plutôt que de s'inquiéter de ce manque de financement, le Sénat s'est concentré sur le financement des fédérations de chasseurs par le contribuable, au prétexte qu'elles exerceraient des missions de préservation de la biodiversité, qui ne sont nulle part définies. Enfin, nous regrettons l'entêtement d'une majorité de nos collègues à faire de ce texte un projet de loi sur la chasse : transformation de l'Office français de la biodiversité en Office français de la biodiversité et de la chasse, sanctuarisation de la chasse à la glu, extension de la période de chasse des oiseaux migrateurs, limitation de l'obligation de collecte des données sur les prélèvements- entre autres mesures. Nous ne pouvons donc pas voter

J'espère qu'elle sortira de notre assemblée en ayant une meilleure image que celle que certains ont peut-être voulu lui inculquer. Absolument ! Pour notre part, nous sommes très satisfaits de la manière dont vous avez eu à coeur que les choses se passent bien, madame la secrétaire

de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.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

commission, l'ensemble du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande